Ce texte témoigne de la priorité qu'accordent le Gouvernement et le Parlement aux petites retraites. Il résulte de l'engagement constant du président André Chassaigne, auquel j'adresse un salut républicain. Permettez-moi de remercier le groupe communiste républicain citoyen et écologiste de l'avoir inscrit à son ordre du jour et de saluer chaleureusement mon collègue Julien Denormandie, ministre de l'agriculture et de l'alimentation, que je sais également investi sur cette question. Ce texte est aussi et surtout le reflet d'un véritable consensus républicain en faveur de la revalorisation des retraites agricoles.

ce consensus s'est de nouveau traduit par l'adoption, à l'unanimité, de la présente proposition de loi par l'Assemblée nationale. Venons-en désormais au contenu de cette proposition de loi. Le texte adopté le 17 juin dernier est très équilibré. Il répond à trois principes que j'estime fondamentaux pour faire prévaloir la justice et la pérennité de notre système de retraite,

un minimum de pension unifié, sans distinction de l'activité professionnelle- exploitant agricole ou conjoint collaborateur. Je rappelle que tel est déjà le cas pour le minimum de pension des salariés. Le deuxième principe respecté dans ce texte est celui de la contributivité. Il est justifié, et même légitime, qu'un exploitant agricole qui a davantage cotisé que son conjoint collaborateur perçoive une retraite complémentaire supérieure et puisse, d'ailleurs, d'ailleurs, en faire bénéficier son conjoint ou sa conjointe, par un niveau de vie commun plus élevé. C'est la raison pour laquelle nous ne souhaitons pas, madame la rapporteure, le rétablissement de l'article 2. 2. Dans un système par répartition fondé, par nature, sur une logique assurantielle, la faiblesse des cotisations de certaines professions se traduit mécaniquement par une pension insuffisante. C'est pourquoi l'article 3 est essentiel à mes yeux. En limitant la durée du statut de conjoint collaborateur à cinq ans, on incite au travail sous des formes rémunératrices- conjoint associé ou salarié -et donc davantage créatrices de droits sociaux. Sans ignorer la communauté de vie des conjoints, cette approche est très importante pour reconnaître le travail de chacun à sa juste valeur. Elle se déploiera progressivement et sera dupliquée pour les artisans et commerçants après la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Lorsque ce dernier prend la forme de la solidarité nationale, cela implique, bien entendu, un prélèvement acquitté par le contribuable. La gratuité n'est donc qu'une apparence. Elle est légitime, dans une certaine mesure, pour tenir compte des aléas de la vie auxquels nous pouvons, toutes et tous, à un moment donné, être exposés. Elle ne saurait toutefois constituer le principe général régissant le financement des droits à retraite. Si nous ne souhaitons pas que le financement de ces droits nouveaux repose sur le coût du travail via une hausse des cotisations, il nous faudra, à terme, repenser le financement de notre protection sociale pour en assurer la pérennité. Mais je crois que ce n'est pas là le débat du jour

L'ensemble des services sont déjà mobilisés pour assurer la bonne mise en oeuvre de la loi « Chassaigne 1 » et permettre le versement de l'indemnité inflation aux retraités éligibles d'ici à la fin

au plus vite. Je vous l'indique clairement : les droits ouverts le seront bien au titre des périodes courant à partir du 1 janvier prochain. conclure mon propos sans faire référence à l'entrée en vigueur de la première loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles les plus faibles, celles des chefs d'exploitation. Coïncidence heureuse du calendrier, c'est aujourd'hui qu'intervient de la manière la plus concrète possible la revalorisation à 85 % du SMIC net agricole, prévue par la loi adoptée en juillet 2020. Ces effets commencent à être visibles, depuis ce matin, sur les comptes en banque des retraités bénéficiaires. Ce sont ainsi plus de 200 000 agriculteurs qui bénéficient d'une hausse de pension de 102 euros par mois

souvent André Chassaigne, cette première proposition de loi représente une avancée majeure pour la reconnaissance à l'endroit de celles et ceux qui n'ont jamais cessé de nous nourrir. Si le texte qui vous est présenté est adopté en l'état, une revalorisation tout aussi importante sera alors possible pour les conjoints collaborateurs. Ces conjoints collaborateurs, pour la plupart- disons-le -conjointes collaboratrices, sont souvent les épouses des bénéficiaires de la première loi. Les différentes mesures envisagées permettront non seulement de se prémunir à l'avenir contre les petites pensions, mais aussi de revaloriser les pensions de plus de 200 000 personnes actuellement retraitées. Pour les femmes qui ont été conjointes collaboratrices toute leur vie, le gain moyen sera de 100 euros par mois.

Permettre à chacun, indépendamment de son activité, de percevoir une pension totale de 1 000 euros pour une carrière complète est d'ailleurs l'un des objectifs qui ont été clairement rappelés par le Président de la République, lors de son allocution du 9 novembre dernier. Soyons donc fiers, madame la rapporteure, madame la présidente de la commission, mesdames, messieurs les sénateurs, de l'avancée significative que nous pourrons accomplir aujourd'hui- je l'espère -par votre vote, sans perdre de vue l'ambition plus large d'un travail rémunérateur et créateur de droits pour toutes et pour tous.

il y a un an et demi, notre assemblée adoptait la proposition de loi Chassaigne, devenue la loi du 3 juillet 2020, qui a permis, depuis le mois dernier, de porter la pension de retraite des exploitants agricoles à 85 % du SMIC pour une carrière complète, soit 1 035 euros par mois. Je tiens d'abord et avant tout à saluer la détermination et la persévérance d'André Chassaigne, qui n'a jamais ménagé ses efforts pour sortir de la misère ceux que la vie n'a pas épargnés. Au nom du groupe CRCE, mais aussi- je crois pouvoir le dire -en notre nom à tous, je lui adresse des remerciements appuyés.

les organisations syndicales du secteur agricole, je vous propose donc de nous contenter des mesures ayant fait consensus à l'Assemblée nationale, qui constituent déjà une avancée. Le groupe CRCE ne manquera pas de proposer d'y revenir à l'avenir. Dans le monde agricole, nombre de conjoints et de membres de la famille apportent, sous diverses formes, leur concours à la gestion des exploitations, sans percevoir de rémunération en contrepartie. Jusqu'en 1999, le conjoint d'un exploitant agricole qui n'était pas déjà affilié à un régime de retraite au titre de son activité professionnelle était, sauf preuve contraire, présumé participer à la mise en valeur de l'exploitation. Cette présomption emportait de manière subie l'application du statut de conjoint participant aux travaux. Les garanties de protection sociale prévues par ce statut étaient, en outre, particulièrement limitées, notamment en matière d'assurance vieillesse. En effet, au-delà de la pension de retraite forfaitaire, le conjoint participant aux travaux ne percevait une pension de retraite proportionnelle que si le ménage avait opté pour un partage à parts égales des points de retraite acquis par le chef d'exploitation. C'est la raison pour laquelle la loi d'orientation agricole de 1999 a créé le statut de conjoint collaborateur. Ce statut revêt un caractère optionnel et permet aux conjoints concernés, à 78 % des femmes, de bénéficier d'une couverture sociale multirisque, incluant une pension de retraite proportionnelle de droit, en contrepartie du versement, par le chef d'exploitation, de faibles montants de cotisations sociales. Le statut de conjoint participant aux travaux a, quant à lui, disparu en 2009. Les autres membres de la famille âgés de plus de 16 ans vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et y exerçant une activité non salariée peuvent exercer en qualité d'aide familial et bénéficient des mêmes garanties. Les statuts de conjoint collaborateur et d'aide familial

Néanmoins, ces statuts produisent aujourd'hui des effets contraires à la noble ambition qui a présidé à leur création et sont devenus de véritables « trappes à faibles pensions ». En effet, afin de ne pas faire peser une charge excessive sur les chefs d'exploitation, qui en sont redevables, les cotisations versées au titre de l'activité des conjoints collaborateurs et des aides familiaux sont fixées forfaitairement sur des assiettes extrêmement faibles, tandis que les cotisations personnelles des chefs d'exploitation sont proportionnelles à leurs revenus professionnels, avec des assiettes minimales plus élevées. Ce différentiel de cotisations n'est pas sans conséquence sur le niveau des pensions servies et, notamment, sur l'accès aux minima de pension du régime des non-salariés En effet, les femmes monopensionnées ayant effectué une carrière complète sous le statut de conjoint collaborateur perçoivent en moyenne une pension de droit direct de 570 euros par mois. Notons toutefois que les polypensionnées justifiant d'une carrière complète parviennent à atteindre 1 017 euros par mois. Le statut de conjoint collaborateur est, d'ailleurs, en déclin : il ne concerne plus que 22 800 personnes à ce jour, soit deux fois moins qu'il y a dix ans et quatre fois moins qu'il y a trente Les pensions servies aux conjoints collaborateurs et aux aides familiaux retraités sont d'autant plus faibles que ces assurés n'ont pas accès aux mêmes minima de pension que les chefs d'exploitation. Tandis que le montant du minimum de pension de base pour une carrière complète, la pension majorée de référence (PMR), diffère selon le statut professionnel de l'assuré, les conjoints collaborateurs et les aides familiaux n'ont pas accès à la garantie de pension à 85 % du SMIC, dont bénéficient les chefs d'exploitation via le complément différentiel de points de retraite complémentaire (CDRCO). Cette différence de traitement, qui se fonde sur le différentiel de cotisations, n'est plus justifiée aujourd'hui, au regard de l'impératif de lutte contre la pauvreté. Par ailleurs, je tiens à souligner que le minimum contributif (MICO) servi par le régime général aux assurés ayant cotisé sur de faibles salaires durant leur carrière, qui constitue le pendant des minima de pension des régimes agricoles, ne varie pas selon la rémunération antérieure. De plus, le non-recours à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) constitue un problème persistant.

à 50 % des bénéficiaires potentiels, proportion qui pourrait se révéler plus élevée encore dans le monde agricole. En effet, les modalités d'attribution et de récupération sur succession de cette allocation, qui s'élevait à 907 euros par mois en 2021, semblent encore largement méconnues. Nombre d'agriculteurs ignorent en effet que l'ASPA n'est récupérée que si l'actif net successoral excède 39 000 euros dans l'Hexagone et 100 000 euros dans les outre-mer, que le capital d'exploitation agricole et les bâtiments indissociables en sont exclus et que le montant des sommes pouvant faire l'objet d'un recouvrement est plafonné annuellement. La proposition de loi qui vous est présentée ce matin apporte des solutions concrètes à ces enjeux majeurs. L'ensemble des mesures qu'elle prévoit concerneraient, en 2022, quelque 214 000 pensionnés, dont 67 % de femmes. Son adoption permettrait d'accroître de 100 euros en moyenne par mois la pension des 70 000 femmes ayant accompli toute leur carrière en qualité de conjoint collaborateur. Elle tend en effet à relever la pension majorée de référence des conjoints collaborateurs et des aides familiaux au niveau de celle des chefs d'exploitation, soit à 699 euros contre 555 euros aujourd'hui. Cette seule mesure, qui concernerait autant le stock de retraités que le flux de nouveaux pensionnés, bénéficierait à 175 000 personnes, dont le gain moyen s'élèverait à 62 euros par mois et, notamment, à 75 euros par mois pour les femmes. De plus, lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a pris l'engagement d'aligner le montant de la nouvelle pension majorée de référence unique sur celui du MICO majoré, soit 705 euros par mois. J'espère que cet engagement sera confirmé. Enfin, le seuil d'écrêtement de la pension majorée de référence, c'est-à-dire le niveau global de pension au-delà duquel la majoration servie est réduite à due concurrence du dépassement, serait fixé au niveau de l'ASPA et passerait donc de 875 euros à 907 euros par mois. Cette mesure bénéficierait à 43 000 personnes. Il s'agit, d'abord, du renforcement de l'information des assurés au sujet des conditions d'attribution et de récupération sur succession de l'ASPA, qui interviendrait non seulement au moment de la liquidation de la pension, mais également l'année précédant l'âge d'éligibilité à l'ASPA, fixé à 65 ans. Ensuite, la possibilité d'exercer sous le statut de conjoint collaborateur serait limitée à cinq ans, comme c'est le cas pour les aides familiaux depuis 2005, de façon à orienter les intéressés vers une activité rémunératrice leur permettant de bénéficier d'une meilleure collègues, j'attire votre attention sur le financement de cette proposition de loi. André Chassaigne proposait la création d'une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières au taux de 0,1 %, qui aurait permis de dégager 450 millions d'euros de recettes. Cette proposition a été rejetée par l'Assemblée nationale avec, évidemment, l'aval du Gouvernement. Or le coût de la revalorisation des pensions devrait entraîner, en 2022, un déficit de l'ordre de 94 millions d'euros. Malgré les lacunes importantes du texte issu de l'Assemblée nationale, l'ensemble des acteurs du monde agricole estiment nécessaire de permettre, sans plus tarder, la mise en oeuvre des mesures ayant fait consensus dès le 1 janvier prochain. La commission partage pleinement cette opinion. Aussi vous propose-t-elle d'adopter cette proposition de loi sans modification. En votant en faveur de ce texte, nous rendrons à nos agriculteurs l'hommage qu'ils méritent. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le 1 novembre 2021 est entrée en vigueur la loi « Chassaigne 1 », qui porte la pension de retraite des chefs d'exploitation de 75 % à 85 % du SMIC. Grâce à la mobilisation des organisations syndicales et à la pugnacité de notre collègue député communiste André Chassaigne, 230 000 actuels et futurs retraités agricoles ont vu leur retraite passer de 914 euros à 1 036 euros net par mois, soit une augmentation d'environ 122 euros net par mois depuis le 1novembre 2021, pour une carrière agricole complète.

En effet, lors de la discussion de la première proposition de loi, l'angle mort des conjoints collaborateurs des exploitants agricoles avait été largement relevé. Notre collègue André Chassaigne a donc remis l'ouvrage sur le métier pour y remédier.

visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles les plus faibles, désormais appelée loi « Chassaigne 2 ». Si la situation de nos agriculteurs demeure difficile face aux lois du marché et à des distributeurs qui ne leur permettent toujours pas de vivre dignement de leur travail, celle des conjoints agricoles et des aides familiaux est encore plus précaire. En effet, le régime des non-salariés agricoles opère une distinction entre les exploitants, qui bénéficient d'une pension minimale de 700 euros pour une carrière complète et les conjoints collaborateurs et aides familiaux, dont la pension s'élève seulement à 555,50 euros. Au 1 janvier 2020, 97 % des retraités relevant du statut de conjoint collaborateur et les deux tiers des retraités aides familiaux étaient des femmes. Ces femmes touchent une pension moyenne de 604 euros par mois si elles ont validé au moins 150 trimestres et de seulement 307 euros par mois quand elles n'ont pas atteint cette durée d'assurance. Cette proposition de loi tend donc à aligner les pensions de référence des aides familiaux et des conjoints collaborateurs sur celles des exploitants agricoles.

Il ne faut pas oublier non plus les 5 000 à 6 000 femmes qui travaillent dans l'exploitation agricole de leur conjoint sans aucun statut. Nous regrettons que les députés La République en Marche aient supprimé du texte la création d'une taxe de 0,1

au-delà des sensibilités politiques, à soutenir cette proposition de loi qui va dans le sens de la justice sociale et d'une reconnaissance du monde agricole dans son ensemble. La parole

J'ai tendance à trouver, en effet, que les lois sont trop nombreuses et trop bavardes. Longtemps, je m'en suis tenue à ce principe. Et puis, un jour, alors que je suis dans la rue, une amie à la retraite, femme de paysan, me téléphone. Soudain, elle fond en larmes : « Il faut faire quelque chose, avec 500 euros par mois, je n'y arrive plus ! instant, tout s'est arrêté. J'étais entièrement concentrée sur cette détresse sincère et humaine, qui m'arrivait d'un petit village de la Nièvre, de la part d'une femme dont je sais qu'elle a travaillé dur, toute sa vie, aux côtés de son époux. J'ai donc déposé une loi. C'était sans savoir que des collègues députés étaient engagés dans la même démarche. J'ai lu dans un journal qu'André Chassaigne, qualifié à juste titre d'« infatigable chantre du monde rural », avait eu le même déclic que moi, quelque temps avant, un jour où un agriculteur lui avait fait un discours sur les retraites agricoles. chacun de vous, dans son cercle amical, local, professionnel, a certainement eu ce déclic. Comment est-il possible qu'après une vie professionnelle physique, continue, éreintante, des femmes et des hommes puissent se retrouver avec d'aussi minuscules retraites ? Que peut-on faire pour eux ?

Le dossier des retraites agricoles en général est en chantier depuis des années. Tout d'abord, la revalorisation de la retraite des chefs d'exploitation, qui atteint enfin 85 % du SMIC ces jours-ci, après un cheminement complexe et tortueux et grâce à la ténacité de notre collègue André Chassaigne. Les conjoints collaborateurs et aides familiaux étaient, jusqu'à maintenant, les grands absents de cette revalorisation tant attendue. Pourtant, il y avait là une urgence humaine et sociale. On ne pouvait pas, décemment, attendre une réforme globale des retraites. On ne pouvait pas accepter que la retraite des chefs d'exploitation augmente enfin quelque peu et que les conjoints, qui sont essentiellement des conjointes et qui ont en général partagé le même quotidien, restent des oubliées,

ont réussi un exercice de haute voltige. En alignant le montant de la pension majorée de référence des conjoints sur celui de la PMR des chefs d'exploitation et en relevant son seuil d'écrêtement, on obtient une augmentation d'environ 100 euros par mois. Je suis extrêmement heureuse et fière de présenter aujourd'hui cette disposition, qui constitue une avancée significative à laquelle je suis très attachée. Sans réserve, le groupe centriste la votera conforme. J'ajoute que, plus que jamais, le moment est bien choisi. Non pas à cause des échéances électorales- si c'est ce que vous avez pu imaginer -, mais à cause de la relance. Car, voyez-vous, quand on perçoit 500 euros par mois, chaque euro de plus ne part pas chez Amazon ou dans de lointains placements. Chaque euro de plus va chez le boulanger du village, chez le livreur de fioul ou chez le garagiste local. Ces euros-là diffuseront dans le tissu fragile de nos petits commerces et artisans ruraux. Ces euros-là constituent notre relance de proximité, celle qui ne peut pas s'échapper et qui sera à 100 % utile, de même que, dans nos communes rurales, un euro de subvention est un euro investi.

Il faudra aller plus loin et cette proposition de loi doit également être un appel. Un appel pour que plus jamais les cotisants et cotisantes agricoles ne se retrouvent, par défaut de cotisations, dans des situations insupportables et indignes. La retraite ne doit plus jamais être une variable d'ajustement. Un appel pour que chacun et chacune se pose, en toute connaissance de cause, la question de son statut dans la durée. Un appel à lutter contre le non-recours à l'ASPA et contre le non-recours aux droits de manière Que nous ayons été plusieurs à défendre ce sujet est une excellente nouvelle ; c'est la preuve qu'il y a là un dossier de première importance. Oui, monsieur le secrétaire d'État, le sujet des petites retraites doit être traité dans sa globalité, mais aujourd'hui, un grand pas est fait. Je vous remercie très sincèrement pour votre engagement sur ce dossier et je remercie les

Les retraites agricoles sont parmi les plus faibles, tous régimes confondus. Le récent rapport des députés Causse et Turquois rappelle en effet que les assurés non salariés et les exploitants agricoles sont surreprésentés parmi les retraités modestes. Au sein du régime des non-salariés agricoles, les conjoints et aides familiaux touchent moins que le minimum vieillesse. Les chiffres sont édifiants : pour une carrière complète, la pension moyenne est de 570 euros par mois, et bien moins encore pour tous ceux ou plutôt, devrais-je dire, toutes celles- il s'agit le plus souvent de femmes -qui n'ont pas cotisé suffisamment. Pour ces dernières, leur opposer un faible effort contributif est indélicat. Comme l'a souligné Mme la rapporteure, le statut de conjoint collaborateur est resté longtemps subi et le partage à parts égales des points de cotisation rarement mis en oeuvre par le chef d'exploitation. Si leur protection sociale s'est régulièrement améliorée depuis 1999, l'article 3 de la proposition de loi visant à limiter à cinq ans la durée d'exercice du statut de conjoint collaborateur leur ouvrira de nouvelles perspectives. du RDSE a d'ailleurs défendu ce dispositif dans le cadre de l'examen du dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je rappellerai aussi que mon groupe est depuis longtemps attentif au sort de l'ensemble des retraités du monde agricole deux de ses anciens membres avaient déposé en 1998 une proposition de loi allant dans le sens d'une nette amélioration de leurs pensions. En tout état de cause, il nous revient à tous ici de réparer cette situation de précarité qui touche des agricultrices dont on sait qu'elles ne ménagent pourtant pas leur peine sur l'exploitation. L'article 1 qui tend à supprimer la prise en compte du statut professionnel pour le calcul du montant de la pension de base minimale apportera davantage d'équité en faveur de ses 175 000 bénéficiaires.

aux conjoints collaborateurs et aux aides familiaux de la garantie d'un revenu minimal de 85 % du SMIC, dispositif que nous avions approuvé l'année dernière à l'unanimité en faveur des chefs d'exploitation. Vous l'avez souvent souligné, monsieur le secrétaire d'État, le coût en serait difficilement supportable. Toutefois, les pistes de financement proposées par le député Chassaigne méritent d'être étudiées pour apporter, à terme, une pierre de plus à l'effort indispensable de revalorisation des petites pensions. Mes chers collègues, en parallèle, nous devons aussi poursuivre le travail de sécurisation des revenus agricoles entamé par la loi dite Égalim. Les retraites agricoles d'aujourd'hui reflètent les revenus tirés de l'agriculture d'hier. Aussi, garantir au plus tôt de meilleurs salaires pour nos agriculteurs est à l'évidence la meilleure façon d'assurer leurs pensions de demain, des pensions qui doivent être le plus dignes possible au regard de leur contribution à la vitalité de nos territoires.

mes chers collègues, je souhaite à mon tour saluer l'examen dans notre hémicycle de cette proposition de loi déposée par André Chassaigne visant à revaloriser les pensions de retraite agricoles des conjoints collaborateurs et des aides familiaux.

puis la première loi Chassaigne du 3 juillet 2020 qui a porté ce montant à 85 % du salaire minimum pour les chefs d'exploitation ayant effectué une carrière complète. dernière disposition s'applique depuis le 1 novembre dernier et les premiers versements à terme échu interviennent donc en ce moment même. Mes chers collègues, nous ne pouvons que nous en réjouir, même si je tiens tout de même à rappeler que cette revalorisation aurait pu s'appliquer trois ans plus tôt, si le Gouvernement n'avait pas choisi en 2018 de la reporter, en ayant recours en séance à la procédure du vote bloqué, alors que le Sénat souhaitait au contraire voter conforme ce texte dès sa première lecture afin de garantir sa mise en oeuvre rapide. Nous espérons donc que l'adoption définitive de cette nouvelle proposition de loi qui concerne les conjoints collaborateurs et les aides familiaux pourra cette fois se dérouler sans encombre, car elle est vivement attendue par l'ensemble des acteurs du monde agricole.

de ce texte instaure une mesure essentielle, en établissant un montant unique de pension majorée de référence, quel que soit le statut de l'assuré non salarié agricole.

Au total, plus de 200 000 personnes pourraient ainsi bénéficier de ces mesures qui représentent une revalorisation de 100 euros par mois en moyenne pour les femmes ayant accompli l'ensemble de leur carrière en tant que conjointes collaboratrices. Cela constitue indéniablement une avancée importante, mais nous ne pouvons que regretter que la majorité de l'Assemblée nationale ait rejeté dans le même temps l'article 2 de la proposition de loi qui élargissait l'application du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire aux conjoints et aides familiaux afin qu'ils puissent bénéficier de la garantie d'un revenu minimal à hauteur de 85 % du SMIC.

Cette information devra être délivrée non seulement au moment de la liquidation de leur retraite, mais également l'année précédant leur éligibilité à cette allocation, ce qui représente une avancée, car l'une des causes du non-recours à l'ASPA pourrait résulter du décalage entre l'âge légal de départ à la retraite, fixé à 62 ans, et celui auquel l'assuré peut solliciter cette allocation, à savoir 65 ans. Nous nous félicitons également que l'article 3 tende à limiter à cinq ans le statut de conjoint collaborateur- cette limitation est déjà applicable aux aides familiaux -afin de les encourager à privilégier un statut socialement protecteur comme celui de coexploitant ou de salarié. Cette disposition a d'ailleurs été étendue à l'ensemble des conjoints collaborateurs, y compris ceux qui seraient déjà en activité lors de la promulgation de la loi. L'article 3 , introduit à l'Assemblée nationale sur l'initiative d'André Chassaigne, prévoit enfin la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur l'application de l'article 9 de la loi Pacte, qui instaure des obligations déclaratives pour les chefs d'exploitation, et sur la situation des conjoints d'agriculteurs dont la situation professionnelle n'est pas déclarée. Au vu de l'ensemble de ces motifs, et malgré nos regrets réitérés quant à la suppression de l'article 2 qui aurait permis de garantir un montant minimal de retraite à 85 % du SMIC aux conjoints collaborateurs et aux aides familiaux, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera ce texte tant il est urgent de confirmer cette première avancée pour se diriger enfin vers des pensions de retraite dignes pour l'ensemble des non-salariés agricoles. La parole

J'ai d'ailleurs une pensée toute particulière pour les 948 exploitations agricoles du département des Yvelines. Céréaliers, maraîchers, éleveurs, primeurs, quel que soit leur domaine, ils démontrent que leur activité évolue afin de préserver la filière. Leur présence est précieuse, car ils assurent un rôle déterminant, notamment dans notre équilibre alimentaire. Comment ne pas rappeler en préambule que la grande majorité des syndicats d'agriculteurs souhaitait la réforme universelle des retraites ? Malheureusement, la covid-19 a contraint le Président de la République à la reporter jusqu'à ce que les conditions économiques et sociales soient réunies. Ces professions ne pouvaient plus attendre. Et il était indispensable de se pencher en urgence sur les pensions du monde agricole, au vu de leur montant. Aussi, c'est bien naturellement que nous avons apporté tout notre soutien à la loi du 3 juillet 2020, rebaptisée Chassaigne 1. de revaloriser les retraites agricoles, portant la pension totale d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en métropole et en outre-mer justifiant d'une carrière complète à 85 % du SMIC net à partir du 1 janvier prochain. Elle concerne 227 000 chefs d'exploitation agricole qui voient leur retraite minimale portée à 1 035 euros par mois. C'est une avancée majeure adoptée avec le soutien du Gouvernement. de loi que nous examinons aujourd'hui complète ces avancées, en améliorant la retraite des collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les anciens conjoints participant aux travaux et les aides familiaux, qui sont à 75 % des femmes. Elle s'inscrit pleinement dans le cadre des travaux conduits par le Gouvernement. Elle s'inscrit également dans la lignée des recommandations de la mission sur les petites retraites confiée aux députés Lionel Causse et Nicolas Turquois par le Premier ministre. Son article 1 prévoit le rapprochement de la pension majorée de retraite et du minimum contributif du régime général. Pour les 175 000 bénéficiaires de cette mesure, le gain moyen s'élèvera à 62 euros par mois et même à 75 euros pour les femmes. L'article 1 prévoit, quant à lui, de renforcer l'information des assurés au sujet des conditions d'attribution et de récupération sur succession de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Le non-recours à l'ASPA est particulièrement élevé dans le secteur agricole en raison des craintes liées à la récupération sur succession des sommes versées. Précisons que cette allocation n'est récupérée que sur la fraction de l'actif net successoral excédant 39 000 euros en métropole et 100 000 euros en outre-mer, tandis que le montant des sommes pouvant faire l'objet d'un recouvrement est plafonné annuellement. Depuis 2011, le capital d'exploitation agricole et les bâtiments indissociables sont même exclus du calcul de l'actif net successoral. L'article 3 tend à limiter à cinq ans la possibilité d'exercer sous le statut de conjoint collaborateur. Cette mesure, vous le rappelez dans votre rapport, madame la rapporteure, fait consensus parmi les organisations syndicales et contribuera à orienter les intéressés vers une activité rémunératrice leur permettant d'acquérir des droits sociaux plus étendus. L'article 3 vient compléter les avancées de la loi Pacte, en clarifiant les obligations de déclaration des conjoints collaborateurs, ainsi que les conséquences d'une éventuelle non-déclaration. Mes chers collègues, le Gouvernement est attaché à trois principes qui ont déterminé sa position dans les débats sur les petites retraites agricoles

lors du discours d'Aurillac, par George Pompidou pour qui l'effort autour de l'agriculture devait nous permettre de « répondre aux besoins de la France et de l'Europe de demain et d'assurer en même temps à nos agriculteurs un niveau de vie convenable Nous l'avons encore bien vu depuis le début de cette pandémie : nos agriculteurs ont sauvegardé notre souveraineté alimentaire. Nous avons parlé en septembre dernier de la question de la rémunération de nos agriculteurs, en examinant la s'agissait de leur assurer un niveau de vie convenable, ce qui n'est pas le cas actuellement. Après une vie de labeur particulièrement intense, la retraite doit apporter de quoi vivre. Je souhaite féliciter le député André Chassaigne pour son engagement constant et reconnu en faveur du secteur de l'agriculture et plus particulièrement des retraites agricoles. Je salue cette proposition de loi qui a le mérite d'apporter une solution à un problème identifié depuis bien longtemps. Lors de son examen, la commission des affaires sociales adopté le texte sans apporter de modification à ses quatre articles. L'entrée en vigueur de plusieurs dispositifs se situant au 1 janvier prochain, nous comprenons l'enjeu. Le sort des conjoints collaborateurs et des aides familiaux est particulier à plusieurs égards : d'abord par leur statut, ensuite par le rôle important qui est le leur au sein d'une exploitation.

comme c'est déjà le cas pour les chefs d'exploitation grâce à la loi Chassaigne 1 de juillet 2020. Cependant, la solution trouvée autour d'un montant unique de pension majorée de référence pour l'ensemble des assurés non salariés agricoles est une avancée

Je souhaite toutefois rappeler que ce manque de cotisation n'est pas volontaire ; il est le résultat du manque de moyens des exploitants, ne leur permettant pas de cotiser suffisamment pour leur conjoint aidant. Autre point essentiel dans cette proposition de loi : la limitation de la durée du statut de conjoint collaborateur. L'encadrement proposé à cinq ans renforce la volonté de protection exprimée dans ce texte. Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, ce texte est une avancée très importante et une question de justice sociale pour les femmes et les hommes qui nous nourrissent. Si les exploitations agricoles fonctionnent, c'est aussi parce que des conjoints collaborateurs et des aides familiaux y déploient un travail continu et de loi apporte des solutions concrètes aux agriculteurs, qui ont travaillé sept jours sur sept et qui, à l'heure de leur retraite, doivent pouvoir eux-mêmes se nourrir et avoir un minimum pour vivre. Le groupe Les Indépendants

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour discuter d'un sujet qui me tient particulièrement à coeur : l'augmentation des pensions de retraite agricoles les plus faibles, pour prendre un peu plus soin de ceux qui nous ont nourris discrètement leur vie durant. Les pensions agricoles d'aujourd'hui sont le reflet de choix historiques posés dans des conditions bien différentes. Elles sont le fruit d'un compromis de l'après-guerre, qui avait choisi d'offrir un régime de retraite à une profession encore très nombreuse participant activement à la reconstruction du pays sans faire peser sur ses revenus des charges sociales trop lourdes. À l'époque, on ne savait pas que les revenus agricoles allaient fluctuer autant ni que la vente des exploitations, censée compléter les revenus des retraités, se compliquerait. Pour le conjoint et les enfants, aucune cotisation- donc aucun droit -n'était prévue, même si ceux-ci participaient aux travaux de l'exploitation leur travail prolongeait celui qui était accompli dans la maison, sans qu'il soit utile de lui associer la moindre reconnaissance d'ordre professionnel. En 1999, les conjoints participant aux travaux de l'exploitation agricole se virent enfin attribuer un statut légal. Ils purent, seulement à partir de 2011, bénéficier d'une retraite complémentaire, mais à des conditions encore moins favorables que les chefs d'exploitation, puisque les cotisations C'est ce qui explique pourquoi, aujourd'hui, les montants moyens des retraites agricoles des non-salariés et des conjoints collaborateurs et aides familiaux sont inférieurs au seuil de pauvreté

Est-ce là notre conception de la justice et de la solidarité nationale pour les quelque 225 000 exploitants, 125 000 conjoints collaborateurs, 204 000 aides familiaux et 390 000 veufs et veuves, dont le travail était vital pour notre pays et qui ne se sont jamais plaints ? Les raisons qui ont conduit à différer continuellement cette revalorisation pourtant si évidente ne sont pas compréhensibles, alors que, dans le même temps, on a consenti d'autres efforts non négligeables pour d'importantes catégories de Français. En fait, on ne devrait même pas débattre de cette question. Je rappelle aussi que la revalorisation des pensions des chefs d'exploitation a déjà pris un certain temps : elle a été adoptée une première fois à l'Assemblée nationale en février 2017 et il a fallu attendre juin 2020, soit près de trois ans et demi, pour que la proposition de loi revalorisant à 85 % du SMIC les retraites des exploitants soit votée, -un report de l'application de cette mesure à novembre de cette année. Je ne suis pas dupe de l'opportunité de ce calendrier, je ne le suis pas non plus en ce qui concerne la présente proposition de loi. Soit ! Ce texte vient donc- à point nommé ... -compléter certains angles morts de la loi de 2020 et rendre en partie justice aux conjoints collaborateurs et aux aides familiaux. Je ne peux que regretter que certaines dispositions proposées par André Chassaigne n'aient pas été conservées lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale et que ne subsiste essentiellement que l'harmonisation de la pension majorée de référence, complétée de l'alignement du plafond d'écrêtement au niveau de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. L'ambition de la proposition de loi initiale était plus décente pour ceux et, surtout, celles qui, au terme d'une vie de labeur et d'astreinte, sont confrontés aux difficultés de la vieillesse et de la dépendance.

et pour le restreindre, en quelque sorte, à un sas de transition dans la profession et sortir d'une logique de couple qui n'est pas sans risque et qui s'ajuste mal avec l'individualisation et l'égalité des droits. Pour aller plus loin, si nous voulions véritablement prendre soin de ceux qui nous nourrissent, il faudrait réfléchir à un régime renouvelé, fondé sur un nouvel équilibre en rapport avec l'actuelle démographie de la profession et le niveau des prix de cession des exploitations. Agir sur les retraites agricoles permettrait de relancer l'attractivité du métier et de réguler le coût de cession des fermes. Même si ce n'est pas l'objet de la discussion de ce jour, ce sont des enjeux que nous ne devons pas perdre de vue.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, après une première loi adoptée en 2020 qui a porté le complément de retraite obligatoire de 75 % à 85 % du SMIC pour les chefs d'exploitation, mesure effective depuis le 1 novembre 2021,

À l'heure où une partie du monde agricole est en crise, où les pratiques sont remises en question, tant d'un point de vue économique qu'environnemental, et où les drames s'accumulent, cette proposition de loi qui vise les plus précaires de la profession est un signe de respect et de compréhension de l'absolue urgence de la situation. Et nous remercions le groupe CRCE de défendre ce sujet. 307 euros : voilà le montant, dans le régime des non-salariés agricoles, d'une pension de conjoint collaborateur ou de conjointe collaboratrice. Ce montant est dérisoire au regard du travail réellement accompli dans l'exploitation Le mécanisme retenu à l'article 1 de ce texte pour revaloriser ces pensions consiste à aligner la pension majorée de référence des conjoints collaborateurs et des aides familiaux sur celle des exploitants. Cela devrait bénéficier à 175 000 pensionnés pour un gain mensuel moyen de 62 euros. Les 25 % les plus pauvres des non-salariés agricoles obtiendront un gain de 106 euros mensuels et les 5 % les plus précaires de 144 euros mensuels. Nous regrettons toutefois que l'extension aux conjoints collaborateurs et aux aides familiaux du bénéfice de la garantie d'un revenu minimal de 85 % du SMIC ait été supprimée sans proposition de Et nous alertons sur la mesure de l'article 3 qui vise à limiter à cinq ans le statut de conjoint collaborateur d'exploitation à l'image du statut d'aide familial. Si nous comprenons cette stratégie qui est d'en finir avec ces sous-statuts, cela signifie qu'il reste cinq en place une véritable politique de revenus pour les agriculteurs et agricultrices, afin de garantir la pérennité des exploitations. Ces sous-statuts existent toujours, car nombre d'exploitations ne sont pas encore en mesure de s'en passer : la question du revenu est donc primordiale.

La vision libérale qui a conduit à la dérégulation des marchés agricoles européens depuis le début des années 1990 perdure. Or, si nous souhaitons des prix équitables pour les producteurs, donc des revenus dignes, et des prix raisonnables pour les consommateurs, il faut des outils de régulation des marchés, sur le stockage, les prix ou encore les volumes de production. Enfin, nous défendons le fait que les droits annuels soient à l'avenir indexés sur le SMIC horaire comme la cotisation minimum, et non sur les prix. En effet, cette configuration d'indexation est pénalisante, d'autant qu'elle est associée à un allongement de la durée de cotisation pour l'obtention du taux plein. Ce sont là des pistes de travail pour un troisième texte sur cet enjeu essentiel : garantir des conditions de vie plus dignes à l'ensemble de la profession.

Cette histoire, c'est celle qu'ont vécue les femmes de paysans pendant des décennies, c'est celle de la grand-mère de mon épouse, Juliette Ampilhac, née Fuzet. Elle est née en 1920, en Haute-Loire,

une situation difficilement supportable et d'offrir une revalorisation significative aux conjoints collaborateurs et aux aidants familiaux, qui ont oeuvré, souvent dans l'ombre et sans bruit, à l'agriculture de notre pays. Je veux rappeler que cette revalorisation a longtemps été ajournée et que 90 % des 493 000 femmes retraitées du régime des non-salariés agricoles percevant une pension inférieure à 1 000 euros par mois ont été conjoint collaborateur ou aide familial au cours de leur carrière.

Par ailleurs, cet article prévoit le relèvement du seuil d'écrêtement de la pension majorée de référence au niveau du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) pour une personne seule, soit 906,81 euros. De telles dispositions permettront d'améliorer la situation des conjoints collaborateurs et des aides familiaux retraités ; il s'agit de mesures de bon sens très largement attendues dans

des agriculteurs, qui ont été malheureusement trop longtemps laissés pour compte. Je veux aussi exprimer mes regrets vis-à-vis de la position adoptée par la majorité gouvernementale à l'Assemblée nationale : elle n'a eu de cesse de réduire la portée du texte d'André Chassaigne.

Le scrutin est ouvert.

le résultat du scrutin. Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence,

invitant le Gouvernement à relancer une initiative internationale multilatérale visant à la concrétisation d'une solution à deux États et à la reconnaissance d'un État palestinien par la communauté internationale, aux côtés d'Israël pour une paix juste et durable entre les peuples, présentée, en application de l'article

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de résolution que nous soumettons à votre approbation a un objet simple : inviter le gouvernement français, qui va présider le Conseil à compter du 1 janvier, à engager au plus vite une nouvelle initiative internationale multilatérale en vue d'aboutir à la concrétisation d'une solution à deux États passant par la reconnaissance d'un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël. Pourquoi cette initiative ? Et pourquoi maintenant ? Parce que, sans une telle initiative, l'inaction internationale perdurera face à la violence de la colonisation qui continue de se déployer en toute impunité, au mépris de toutes les résolutions de l'ONU votées par la France comme par la grande majorité de la communauté internationale. Parce que, si cette violence perdure, la paix ne viendra jamais, ni pour les Palestiniens ni pour les Israéliens, et ce foyer d'insécurité régionale et internationale Jamais ne sera acceptée l'annexion par Israël des terres destinées à un État palestinien, comme l'a montré en mai dernier la révolte massive de la jeunesse palestinienne dans tous les territoires, y compris en Israël. Cette Cette révolte a envoyé un message au monde entier : la conscience nationale palestinienne est toujours là, debout. Parce que la France, enfin, est la mieux placée pour prendre cette initiative, après le discrédit du prétendu du siècle scellé par l'administration de Donald Trump. Trump. Deux ans après le vote par notre assemblée, et par l'ensemble du Parlement, d'une résolution sur la reconnaissance d'un État de Palestine, à la fin de 2014, la France était, le 15 janvier 2017, à l'initiative d'une rencontre réunissant 70 pays pour relancer une dynamique internationale en faveur d'un processus de règlement politique. C'était, à l'époque, un nouvel espoir. Nous savons qui a brisé l'élan alors suscité : Donald Trump, investi à la tête des États-Unis à peine cinq jours après ce sommet de Paris. de Paris. Il avait annoncé la couleur dès sa campagne électorale ... Dès décembre 2017, malgré la désapprobation internationale, et celle de la France,

Un an plus tard, la Maison-Blanche rétrogradait le niveau de sa représentation diplomatique auprès des Palestiniens, tout en entamant des discussions avec Israël autour de ce que Tel-Aviv et Washington allaient improprement baptiser le du siècle. Cet accord, présenté en janvier 2020 et discuté uniquement avec le gouvernement de Benyamin Netanyahu, était une caricature, visant à enterrer une solution de paix juste et durable. En autorisant l'annexion de la vallée du Jourdain et d'un tiers de la Cisjordanie, en légalisant les colonies du plateau du Golan syrien et de Jérusalem-Est, Washington privait les Palestiniens de 70 % de leurs territoires reconnus dans la limite des frontières de 1967 et d'une future capitale pour leur État. En autorisant l'État d'Israël à créer un statut de résident, aux droits civiques et de circulation limités, pour les Palestiniens installés dans les territoires occupés ou annexés, et en rejetant tout droit au retour des réfugiés palestiniens, il foulait aux pieds, une fois encore, le droit international. Ce plan, largement critiqué par la très grande majorité des États du monde, n'offrait aucune solution crédible. Malheureusement, s'il a, plus que jamais, mené le conflit dans l'impasse, et a été compris par les gouvernements israéliens successifs comme un feu vert donné à l'accélération de l'annexion et de la colonisation, il a aussi conduit l'ensemble des acteurs internationaux, dont la France, à un attentisme coupable : il fallait attendre, toujours attendre, de voir ce que donnerait le plan américain. Aujourd'hui, on a vu et il faut sortir d'urgence de cet immobilisme, qui devient sinon une complicité de fait, malgré nos déclarations officielles, avec la politique d'annexion L'élection de Joe Biden a tourné une page, dans la mesure où le plan Trump n'est plus la feuille de route officielle de l'administration américaine. Mais tout le monde sait que l'administration Biden ne prendra pas d'elle-même, pour le moment, d'initiative majeure. C'est pourquoi la France doit le faire, comme elle l'avait fait en 2017. C'est ce que le ministre palestinien des affaires étrangères et la nouvelle ambassadrice de Palestine en France sont venus dire à la France lors du Forum de la paix et, ici même, au président du Sénat lors d'une entrevue à l'occasion de ce Forum. La France est attendue. Elle peut jouer un rôle essentiel. Le Sénat, en adoptant cette résolution, peut contribuer à ce déblocage. Car nous ne pouvons détourner le regard. Sur place, la situation est plus dramatique que jamais. Une fois la page Netanyahu tournée, la colonisation repart de plus belle, avec la nouvelle coalition menée par Naftali Bennett. Fervent défenseur de la colonisation et de l'annexion, ce dernier accélère la politique agressive de son prédécesseur. Les enquêteurs dépêchés par l'ONU, mais aussi organisations non gouvernementales présentes dans les territoires palestiniens, attestent tous de cette augmentation des violences, des expulsions, des déplacements forcés et illégaux de populations palestiniennes. palestiniennes. Le rapport de l'organisation non gouvernementale Breaking the Silence paru en juillet dernier est très clair : « Cette violence est un instrument pour s'approprier plus de terres. La frontière est très mince entre les colons, pour certains armés par le ministère de la défense, et les soldats qui, parfois, vivent eux-mêmes dans les colonies ou partagent la même idéologie.

Les violences ont atteint un tel stade que ce sont aujourd'hui la Cour pénale internationale et une commission d'enquête spéciale de l'ONU qui mènent des investigations contre Israël pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et atteintes aux droits humains. Qu'est devenu le projet de David Ben Gourion qui, dans sa déclaration du 14 mai 1948, proclamait : « Israël assurera une complète égalité de droits sociaux et politiques à tous ses citoyens, sans distinction de croyances, de race ou de sexe » Qu'est devenu son appel à la paix, assurant qu'Israël tendait « la main de l'amitié, de la paix et du bon voisinage à tous les États » ? Qu'ont fait les gouvernements Netanyahu et Bennett de la déclaration de Yitzhak Rabin du 4 novembre 1995 : La violence sape les bases de la démocratie israélienne. Elle doit être condamnée et isolée. Ce n'est pas la voie d'Israël. [ ...] Je veux dire sans détour que nous avons trouvé un partenaire pour la paix chez les Palestiniens, l'OLP.

appliquer une souveraineté d'Israël sur les territoires occupés, quadriller et scinder les territoires palestiniens, faire des colonies des banlieues d'où aller rapidement dans les centres économiques, et éviter aux colons la traversée de villages palestiniens. Ce projet, inacceptable pour les Palestiniens, contraire à tous les engagements internationaux et à ceux de la France, hypothèque aussi gravement l'avenir pour les Israéliens. Les colonies ne sont pas viables économiquement, et l'avenir économique d'Israël repose aussi sur le travail de Palestiniens de plus en plus nombreux. Que veut devenir Israël ? Un régime d'apartheid ? Où mène, en fait, ce projet méthodiquement appliqué pour expulser, en toute illégalité, les Palestiniens de territoires que la communauté internationale leur reconnaît ? Lors du débat organisé au Sénat sur notre initiative l'an dernier, l'ensemble de nos groupes, et le Gouvernement, qualifiaient le moment que nous vivions de « tournant historique Historique, car de la réaction internationale au plan Trump dépendraient la crédibilité de nos organisations multilatérales et la viabilité d'une perspective de paix entre Israéliens et Palestiniens.

Les conditions de la réussite ne sont pas encore réunies, nous diront peut-être certains, mais c'est l'inaction qui construit chaque jour le chemin périlleux et indigne vers un point de non-retour qui signifiera inévitablement de nouvelles explosions meurtrières. Nous affirmons tous ici notre attachement à la solution à deux États. Cet attachement doit aujourd'hui se prouver par l'action. Il y va de la crédibilité de notre parole sur la scène internationale,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mes premiers mots sont destinés à la famille de notre collègue Catherine Fournier et à ses proches, pour leur adresser mes plus sincères condoléances. Comme à eux, Catherine va beaucoup nous manquer. Avant de commencer mon propos, monsieur le ministre, j'aimerais revenir sur la visite du Président de la République au Moyen-Orient le week-end dernier. Pendant quarante-huit heures, j'ai eu le privilège de faire partie de la délégation qui a accompagné Emmanuel Macron dans ses visites de travail aux Émirats arabes unis, au Qatar et en Arabie Saoudite. Ce voyage fait apparaître des résultats économiques spectaculaires, qui renforceront l'emploi en France ... C'est exact ! ... et la coopération dans la lutte contre le terrorisme s'est accrue. L'annonce opportune de la démission du ministre de l'information libanais, la veille de l'arrivée du Président de la République en Arabie Saoudite, a permis de débloquer la situation à Djeddah et de repartir de l'avant pour oeuvrer en faveur de la stabilité régionale. Nous nous réjouissons d'observer une France qui gagne la France a retrouvé son statut international de force d'équilibre face aux grandes puissances. Vous avez raison ! Ce succès est à mettre au crédit du Président de la République et de notre diplomatie, que je souhaite ici saluer. À l'heure où le Parti communiste chinois viole les droits de l'homme à l'échelle industrielle en République populaire de Chine et à Hong Kong ; au moment où le gouvernement communiste chinois mène une campagne brutale de persécution contre les Ouïghours, en se livrant à des abus qui comprennent l'internement d'au moins un million de personnes, le travail forcé généralisé et la stérilisation forcée de masse ; alors que de nouvelles preuves révèlent le rôle du président Xi Jinping et d'autres hauts responsables du gouvernement communiste chinois dans la mise en place de politiques répressives dans la région ouïghoure, ouïghoure, le groupe communiste du Sénat préfère nous faire débattre dans l'urgence du conflit israélo-palestinien ! La proposition de résolution sur laquelle nous débattons aujourd'hui intervient à une date anniversaire charnière dans l'histoire du dialogue israélo-palestinien. Il y a trente ans, l'année 1991 marquait à bien des égards un bouleversement dans l'ordre mondial. Année de deuil pour les communistes, elle s'est soldée par la démission, le 25 décembre 1991, du président de l'URSS, Mikhaïl Gorbatchev, marquant la fin supposée de l'histoire. Surtout, cette année 1991 s'est révélée être le début d'une nouvelle ère, où les conflits qui couvaient dans le monde depuis des décennies, et particulièrement au Moyen-Orient, ont depuis éclaté. En parallèle de la guerre du Golfe, nous assistions aux prémices d'interminables négociations entre Israël et les territoires palestiniens occupés, mais aussi entre Israël et l'ensemble des pays arabes voisins, pour la normalisation de leurs relations. Avec la conférence de Madrid en 1991, la diplomatie établissait un véritable pas en avant dans la résolution du conflit israélo-palestinien. Les nombreuses réunions à Oslo qui s'ensuivirent ont permis de poser les jalons pour la déclaration de principes signée à Washington le 13 septembre 1993 et symbolisée par la poignée de main historique entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. Il s'agissait là du premier des accords d'Oslo, qui leur valut le prix Nobel de la Paix, en compagnie de Shimon Peres. Ces accords contenaient les principes généraux régissant l'administration autonome palestinienne, sur une période transitoire de cinq ans. La déclaration contenait aussi un accord général visant à transférer progressivement aux Palestiniens la responsabilité civile et politique sur la bande de Gaza et la Cisjordanie, et à leur permettre de gérer leurs affaires de façon autonome. En définitive, à l'issue de cette période transitoire, l'Autorité palestinienne devait devenir l'embryon d'un État palestinien indépendant. Il n'en a rien été. La violence de la seconde intifada enterrera définitivement le processus d'Oslo. Trente ans après le début des négociations, force est de constater que la résolution du conflit israélo-palestinien est dans une impasse. Pis encore, en dépit des multiples résolutions de l'ONU et des avertissements adressés par la communauté internationale aux protagonistes de ce conflit, ce dernier s'est profondément radicalisé, aggravant chaque jour un peu plus la violence et la haine entre les deux camps. Le 1 décembre dernier, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une série de résolutions invitant à des pourparlers de paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Ces négociations sont indispensables pour parvenir à une solution à deux États, qu'une très grande majorité de pays dans le monde appelle de ses voeux. De nombreux obstacles empêchent malheureusement ce règlement diplomatique du conflit. Chacun reconnaît sur ces travées que la solution à deux États serait la plus louable et permettrait enfin d'instaurer la paix et la stabilité dans la région. Pour autant, les conditions du dialogue entre les protagonistes ne sont aujourd'hui pas réunies. La position de la France et de l'Union européenne est très claire depuis de nombreuses années. Plusieurs paramètres sont indispensables pour résoudre ce conflit, à savoir des frontières fondées sur les lignes du 4 juin 1967, avec des échanges agréés de territoires équivalents ; des arrangements de sécurité préservant la souveraineté du futur État palestinien et garantissant la sécurité d'Israël une solution juste, équitable et agréée au problème des réfugiés ; enfin, un arrangement faisant de Jérusalem la capitale des deux États. C'est dans cette optique que la France et l'Union européenne doivent être en mesure de jouer un rôle moteur dans la résolution de ce conflit, qui est désormais interdépendant avec les crises qui se multiplient dans la région. Notre groupe souhaite indiquer que cette proposition de résolution n'est pas l'outil le plus pertinent pour faire avancer la paix au Moyen-Orient. En faisant porter la responsabilité de la situation à Israël et aux États-Unis, le vote d'aujourd'hui incite davantage à la division et sera susceptible de surinterprétations plutôt qu'il ne constituera un appel à l'unité et au dialogue.

Force est de constater que la reconnaissance de l'État de Palestine par 135 États dans le monde n'a pas réglé la question du conflit israélo-palestinien, loin de là. L'inscription de ce texte à l'ordre du jour, à peine une semaine avant son examen en séance publique, n'a pas permis d'échanges concertés et sereins sur la question, ce que je déplore. Je ne peux m'empêcher de penser que la décision du groupe communiste d'inscrire à la va-vite cette résolution à son ordre du jour réservé apparaît comme une exploitation politicienne du malheur d'un peuple et servira des intérêts de politique nationale, à seulement quelques mois d'une élection présidentielle. Ce comportement nous attriste et nous sommes plusieurs à considérer qu'il n'est pas à la hauteur de la vision et des travaux du Sénat ni de l'engagement de nos illustres prédécesseurs. Cette proposition de résolution constitue donc un voeu pieux, qui se heurtera au mur des réalités. Le groupe Union Centriste votera dans sa majorité contre ce texte. En ce qui me concerne, je ne prendrai pas part au vote. Le débat impose que chacun écoute,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de résolution que nous étudions aujourd'hui renvoie à un conflit s'étirant depuis plusieurs décennies. Entre tensions, promesses de paix déçues, déstabilisations et escalades, le conflit israélo-palestinien semble être sans fin. Relancer dans notre assemblée la question palestinienne, mes chers collègues, c'est surtout relancer la question suivante : si une solution à deux États est souhaitable dans l'absolu, est-elle toujours viable ?

Les efforts diplomatiques se sont ensuite poursuivis, avec la conférence de Madrid en 1991, les accords d'Oslo en 1993, le sommet de Camp David en 2000, ou encore la conférence d'Annapolis en 2007. Toutes ces rencontres se sont soldées par l'échec de l'instauration et de la pérennisation d'une solution à deux États. Il est nécessaire de revenir sur deux points particuliers pour tenter de comprendre l'origine de ces faillites diplomatiques à répétition. Ces deux points, à mon sens, expliquent également en partie la stagnation actuelle des négociations. D'une part, la Palestine souffre d'un certain déficit démocratique, dans la mesure où les dernières élections législatives remontent à 2006, et que les élections prévues cette année ont été reportées. Trouver le bon interlocuteur pour entamer un processus de paix est essentiel, et ce dernier doit bénéficier d'une légitimité démocratique incontestable pour que le dialogue diplomatique ne soit D'autre part, une entrave inconditionnelle à la création d'un État palestinien est la multiplication des colonies de civils israéliens, qui morcellent toujours plus le territoire palestinien et la souveraineté du peuple palestinien, et qui réduisent surtout les terres dont disposerait le potentiel État palestinien. Je rappelle que les Nations unies ont fermement condamné l'implantation de ces colonies, dénoncées comme contraires au droit international.

Ces quelques interrogations témoignent de la complexité de la situation israélo-palestinienne, et doivent nous enjoindre de rationaliser le plus possible ce débat afin de ne pas tomber dans le piège des réactions passionnées méconnaissant le caractère clairement non manichéen de cette situation : il n'y a pas les bons, d'un côté, et les mauvais, de l'autre. Il est évident que notre groupe, tout comme cette assemblée, désire une conciliation juste des aspirations nationales israéliennes et palestiniennes, dans le respect des droits de l'homme, et le le retour à la paix dans une région trop longtemps déstabilisée, qui est aussi la matrice d'autres conflits ailleurs dans le monde. La paix n'est pas et ne sera jamais l'exception ! Pour toutes ces raisons, le groupe du RDSE s'abstiendra.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le 29 novembre, lors de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a averti que les violations persistantes des droits des Palestiniens ainsi que l'expansion des colonies israéliennes mettaient en péril la perspective d'une solution à deux États.

Après un cessez-le-feu sans condition préalable entre le Hamas et les forces israéliennes, l'arrêt des hostilités n'a pourtant pas apaisé les tensions à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Tant que les Palestiniens subiront la colonisation et le blocus de Gaza, on ne peut pas s'attendre à une issue favorable. Les violences vont et le silence de l'Europe est assourdissant. Le danger réside aussi dans le fait que nous nous accoutumons aux tourments, aux morts, aux bombardements, au déchirement de ces populations. Cette situation perdure depuis des années, sans le moindre changement significatif.

Depuis le vote de la résolution du Sénat en 2014, qu'a fait la France ? Elle a opté pour une position d'observatrice. Le sujet est inflammable. On préfère donc la passivité, plutôt que d'entamer des pourparlers

Or il y a urgence à agir, car le conflit israélo-palestinien est entré dans une phase critique. Dans quelques semaines, la France prendra la présidence du Conseil de l'Union européenne. C'est l'occasion idéale d'inscrire la paix à l'agenda européen, en proposant la reconnaissance de l'État de Palestine aux côtés de l'État d'Israël. Il est à craindre que la dernière solution ne soit un État binational avec égalité des droits entre Israéliens et Palestiniens

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il y a sept ans, avec émotion, je montais à cette tribune en tant que premier signataire d'une proposition de résolution invitant le gouvernement français à reconnaître l'État de Palestine. Mais, depuis son adoption par le Sénat et l'Assemblée nationale, force est de constater que le processus de paix est au point mort. La France qui, depuis le Brexit, est le seul pays de l'Union européenne à être membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, doit agir pour préserver la solution à deux États, en n'abandonnant ni l'exigence de sécurité pour Israël ni celle de justice pour les Palestiniens. La France a, certes, accueilli une conférence internationale

adoptait une loi légalisant les colonies sauvages en Cisjordanie, au mépris de la résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations unies. Cette loi était déjà un pas vers l'annexion formelle de la Cisjordanie. Le 19 juillet 2018, le parlement israélien adoptait une loi fondamentale disposant qu'Israël est « l'État-nation du peuple juif », avec Jérusalem pour capitale et l'hébreu comme seule langue officielle. Le texte va donc à l'encontre des principes démocratiques et institutionnalise des discriminations raciales envers les Arabes israéliens. Au printemps 2020, Donald Trump dans un plan qu'Israël annexe 30 % de la Cisjordanie, laissant aux Palestiniens un État constitué de plusieurs cantons discontinus et entourés de territoires israéliens, dépourvu de toute souveraineté. Qui mieux que la France peut agir ? La France ne doit pas se résoudre à abandonner l'objectif d'un État palestinien vivant dans la paix et la sécurité au côté de l'État d'Israël au sein de frontières internationalement reconnues et avec Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest pour capitales des deux États. Aussi, en ma qualité de président du groupe d'amitié France-Palestine de notre Haute Assemblée, j'appelle une nouvelle fois solennellement le gouvernement français à reconnaître l'État de Palestine. Reconnaître la Palestine comme un État, ce serait se conformer au droit international. Et lorsqu'on est législateur, on se doit d'être du côté du droit. Au nom du droit inaliénable à l'autodétermination, le peuple palestinien est fondé à se doter d'un État.

C'est aussi l'assurance de la paix et de la sécurité pour Israël ! Il ne se passe pas un jour sans qu'un Palestinien subisse une attaque perpétrée par des colons israéliens.

Selon les estimations israéliennes et palestiniennes, au moins 675 000 Israéliens habitent aujourd'hui

qui puisse être envisagée pour qu'Israéliens et Palestiniens vivent à égalité de droits et de devoirs. Je fais mention de ces échanges pour faire taire la petite musique, que l'on entend parfois, sur la possibilité de la création d'un État unitaire. Je m'oppose absolument à une telle idée, car je pense qu'elle relève du mythe et n'a aucune chance de se réaliser. Mes chers collègues, que la solution à deux États n'ait pas encore abouti ne signifie nullement que ce n'est pas la bonne cela signifie simplement que nous avons échoué jusqu'à présent à la mettre en oeuvre quoi qu'il en coûte. Car, pendant pendant ce temps, des millions de Palestiniens continuent d'être privés de leurs droits fondamentaux et soumis au régime militaire. Durant les sept décennies d'existence d'Israël, il n'y a eu que de six mois pendant lesquels les Palestiniens n'ont pas été placés sous l'autorité d'un gouvernement militaire étranger qui confisque leurs terres. Depuis dix ans que je préside le groupe d'amitié France-Palestine, je rappelle mon attachement à la solution à deux États et ma volonté de voir enfin la Palestine reconnue. Que faut-il faire ? Je continue de penser qu'il n'y a pas d'autre démarche possible que la reconnaissance de l'État de Palestine. Elle doit même être pour moi un préalable à l'organisation de toute conférence internationale. Ne pas reconnaître la Palestine comme État, c'est accepter que la situation actuelle perdure et que les peuples palestinien et israélien continuent à vivre dans un climat de violence

trop importants. Le Gouvernement français doit agir, et il doit le faire maintenant. Aussi, je soutiens pleinement la proposition de relancer

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette dernière année, la situation sécuritaire à Gaza est demeurée hautement instable, rythmée par des incidents récurrents opposant Israéliens et Palestiniens et des annonces, de la part des autorités israéliennes, de constructions de nouveaux logements dans les colonies de Cisjordanie et de Jérusalem-Est qui ont alimenté les tensions. Dans le contexte de la future présidence française du Conseil de l'Union européenne, cette proposition de résolution « invite le Gouvernement à engager, au niveau européen et international, une initiative internationale en vue d'aboutir à la concrétisation d'une solution à deux États et à la reconnaissance d'un État palestinien par la communauté internationale, aux côtés d'Israël pour une paix juste et durable entre les deux peuples Elle justifie cette demande par « l'aggravation des atteintes aux droits, reconnus par l'Organisation des Nations unies, des Palestiniens par l'État d'Israël », « les multiples condamnations internationales dont a fait l'objet l'État d'Israël, notamment au sujet de la colonisation et l'occupation de territoires palestiniens », « le blocage actuel des discussions malgré l'initiative prise par la France en 2017 », puis le plan de paix « malvenu et déséquilibré » de Donald Trump. Les conditions d'un règlement du conflit israélo-palestinien reposent sur trois principes : le droit international et les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, avec dernièrement la résolution 2334 l'établissement de deux États indépendants, démocratiques, viables, avec Jérusalem comme capitale des deux États, souverains dans des frontières sûres et internationalement reconnues sur la base des lignes du 4 juin 1967 celle de la négociation directe entre Palestiniens et Israéliens, et non une décision unilatérale. Le groupe RDPI soutient la position constante de la France, portée par les voix du Président de la République, Emmanuel Macron, et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. La France appelle les deux parties à revenir négocier de bonne foi et à arrêter les prises de décisions unilatérales illégales et les actes de violence. La France condamne sans ambiguïté les tirs de roquettes depuis Gaza vers les zones habitées d'Israël, qui constituent également des violations du droit international. Paris a un engagement indéfectible en faveur de la sécurité d'Israël. La France rappelle régulièrement que la politique israélienne de colonisation dans les territoires palestiniens occupés est illégale au regard du droit international et condamne systématiquement les décisions des autorités israéliennes de construire de nouveaux logements en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. viens à l'esplanade des mosquées : il existe un historique, internationalement acté, qui doit être préservé strictement. La Jordanie joue un rôle spécifique sur les lieux saints de Jérusalem. L'annexion ne serait donc dans l'intérêt ni des Israéliens, ni des Palestiniens, ni des Européens, ni de la communauté internationale, qui ont investi beaucoup d'efforts diplomatiques pour la résolution du conflit. Par ailleurs, la France contribue activement à la réponse humanitaire dans les territoires palestiniens, avec 2,2 millions d'euros en 2020, grâce à plusieurs projets financés par le centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des affaires étrangères auprès d'ONG humanitaires opérant dans l'ensemble des territoires palestiniens. Afin d'appuyer les efforts de l'Autorité palestinienne dans la lutte contre la pandémie, la France a apporté une aide de près de 3 millions d'euros en 2020 par le biais de l'Agence française de développement. La France soutient aussi les activités du comité international de la Croix-Rouge dans ces territoires. À ces montants consacrés à l'aide humanitaire, s'ajoute l'aide budgétaire française apportée à l'Autorité palestinienne, soit 16 millions d'euros en 2020. Ces financements se sont poursuivis en 2021, et ils ne s'arrêteront pas en 2022. Nous nous en félicitons. Nous formons le voeu qu'une paix durable puisse être atteinte au Proche-Orient. Pour que ce voeu puisse être pleinement réalisé, plusieurs attentes pourraient être satisfaites des deux côtés. Nous partageons l'avis que le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a émis avant-hier devant notre commission des affaires étrangères, appelant les acteurs à rétablir avant tout la confiance entre eux, en remédiant à tout handicap qui empêche actuellement le processus de paix de reprendre pleinement. Pour aboutir à deux États, il faut d'abord que des mesures de confiance soient mises en oeuvre. Pour le moment, les conditions ne sont pas pleinement réunies. Nous constatons avec regret que plusieurs pas en arrière ont été effectués. Du côté d'Israël, on peut désormais espérer que la proportionnalité des réponses et la stabilité de la zone soient assurées et que son gouvernement arrête les décisions de colonisations illégales à petits pas, car elles alimentent grandement les tensions. Du côté palestinien, la fixation d'un calendrier électoral et d'une date d'élections précise pourrait être un facteur stabilisant. La population en est demandeuse, et cette demande est plus que légitime. Nous appelons de nos voeux qu'Israël garantisse impérativement la tenue de ces élections dans Jérusalem-Est. Nous formons l'espoir que les travaux du format d'Amman avec, autour de la table, la Jordanie, l'Allemagne, l'Égypte et la France se poursuivent et puissent aboutir à une relance des négociations. Mentionner d'emblée, dans les conditions que je viens d'évoquer, sur un pied d'égalité la solution à deux États et la reconnaissance de la Palestine consiste à assimiler une chose à l'autre. l'autre. Ce serait une provocation finalement assez peu opportune. La situation sur place s'enflamme tellement vite qu'il serait maladroit de s'immiscer aujourd'hui dans cet équilibre précaire trouvé à la suite du cessez-le-feu mettant fin aux violences de mai dernier,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui nous rappelle que le conflit israélo-palestinien n'est toujours pas réglé et fait encore de nombreuses victimes. Peu après la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, alors que la situation est déjà difficile en Palestine entre Juifs et Palestiniens, les Britanniques se dessaisissent de leur mandat au profit de Afin de mettre un terme aux tensions, l'ONU propose en 1947 un plan de partage de la Palestine. Les instances israéliennes l'approuvent, mais les Palestiniens le rejettent. Le conflit qui s'est ensuivi fait encore l'objet d'une attention particulière de la communauté internationale. Une résolution pérenne de cet affrontement implique nécessairement un accord politique et le respect des deux peuples. La solution proposée par la communauté internationale, conforme au droit international, consiste en la coexistence de deux États, l'un palestinien, l'autre israélien. Le 29 novembre dernier marquait le soixante-quatorzième anniversaire du plan de partage décidé par les Nations unies. En cette Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, António Gutteres, secrétaire général de l'ONU, a dénoncé les violations des droits des Palestiniens. Il a en outre mis en garde contre l'expansion des colonies israéliennes en rappelant que celle-ci met en péril la solution à deux États. Ces annonces n'ont évidemment pas été favorablement accueillies par Israël, qui continue aussi de subir des attaques du Hamas.

L'ONU n'est pas parvenue à apporter la paix. Ses résolutions restent lettre morte, et les acteurs concernés privilégient leurs intérêts immédiats aux dépens du droit international et de leurs intérêts à long terme. Nous avons vu le président Trump proposer un nouveau plan de partage et reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël au mépris de la décision prise par l'ONU. Le multilatéralisme s'en est trouvé affaibli. La solution à deux États est la seule que nous devons défendre, parce qu'elle est la seule qui respecte le droit des peuples, donc la seule capable d'aboutir à une paix durable. La sanctuarisation de deux États doit apporter la sécurité pour Israël et la Palestine, afin de leur permettre de vivre en paix. La diplomatie française n'a jamais cessé d'oeuvrer en faveur de la solution à deux États. Il ne nous paraît pas opportun d'inviter le Gouvernement à privilégier un mode d'action plutôt qu'un autre. Nous voyons les relations diplomatiques au Moyen-Orient évoluer. La France soutient la solution à deux États dès qu'elle en a l'occasion, tant à la tribune de l'ONU que dans certaines de ses relations avec les pays du Moyen-Orient. Le 7 décembre dernier, la France et le Qatar ont ainsi publié un communiqué de presse conjoint rappelant leur attachement à la solution à deux États. Nous souhaitons qu'elle aboutisse avec, bien entendu, une reconnaissance mutuelle nécessaire apportant la sécurité aux deux peuples. Notre groupe soutient donc la décision de l'ONU, mais cela doit être reproposé par la France et l'Union européenne au moment le plus

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, par cette proposition de résolution en faveur de la reconnaissance d'un État palestinien par la communauté internationale, nos collègues du groupe communiste entendent inviter le Gouvernement à engager une initiative internationale en vue d'aboutir « à la concrétisation d'une solution à deux États et à la pour une paix juste et durable entre les deux peuples ». Est-il besoin de rappeler que la position constante de la France repose précisément sur l'établissement de deux États vivant côte à côte dans les frontières reconnues et établies sur les lignes du 4 juin 1967, avec pour l'un et l'autre Jérusalem pour capitale Est-il besoin de rappeler encore que nous sommes tous favorables à la solution à deux États ? Ce processus est en principe acceptable par l'État d'Israël comme par la Palestine. Alors quel est le sens d'une « énième » proposition de résolution ? Rappelons-nous l'initiative de notre collègue Gilbert Roger, qui avait présenté en 2014 une proposition de résolution invitant la France à reconnaître l'État palestinien. À l'époque, Christian Cambon avait très justement mis en garde sur la signification de nos actes : reconnaître un État de façon symbolique n'est qu'une reconnaissance de « papier » ; ce n'est pas reconnaître un État à part entière. Nous avions donc voté contre. Et nous avions raison, car la reconnaissance unilatérale, fût-elle celle de la France, n'est pas en soi un instrument de la paix et ne lève aucun des obstacles qui ont rendu impossible cette reconnaissance jusqu'à présent. En tout cas, c'est un constat que nous pouvons faire collectivement sans qu'il soit compris comme une critique envers les auteurs de la proposition de résolution. Un processus est en cours, et il ne peut passer que passer que par une reconnaissance mutuelle fondée sur la paix et la sécurité. La paix au Proche-Orient ne peut reposer que sur une logique multilatérale associant nos partenaires européens et arabes. Oui, la donne géopolitique a changé. Avec la signature des « accords d'Abraham », les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Maroc et le Soudan ont reconnu l'État d'Israël. C'est un encouragement pour recréer la confiance. Mais la crise de Gaza du mois de mai dernier entre Israël et le Hamas nous montre aussi toute la fragilité de l'exercice. D'une part, l'Autorité palestinienne rencontre une crise de légitimité. D'autre part, malgré des signes d'ouverture, la plateforme politique du nouveau gouvernement israélien ne s'engage pas officiellement dans la reprise des négociations vers la solution à deux États. À cet égard, deux constats doivent être posés. la confiance ne peut pas se tisser sans que cessent les actes terroristes et sans que la sécurité d'Israël soit garantie. Deuxièmement, la poursuite de la colonisation des territoires palestiniens est illégale en droit international. Aussi, la présente proposition de résolution n'apporte pas d'éléments que ne porte déjà notre diplomatie et que ne portera la France à la présidence du Conseil de l'Union européenne. Cette présidence doit certainement être l'occasion de mobiliser nos partenaires européens en faveur d'une reprise du dialogue. Ce processus est à l'oeuvre et doit se poursuivre. Et, là encore, il faut se garder d'un excès d'optimisme

à l'est, du nucléaire iranien, de la Syrie et de l'Irak, du Yémen au sud et de la Libye à l'ouest, ces crises occupent le premier rang des préoccupations. L'attitude des États-Unis laisse les acteurs locaux très interrogatifs après le retrait précipité d'Afghanistan et le basculement des priorités américaines vers la zone indo-pacifique et la Chine. Dans ce concert de nations, il faut réaffirmer que la France est l'amie des Israéliens et l'amie des Palestiniens. Ce n'est pas en prenant fait et cause, comme le fait cette proposition de résolution dans ses considérants, pour l'un des deux amis que nous les conduirons à la table des négociations. Nous devons préserver l'équilibre de la position de la diplomatie française, qui doit continuer à maintenir une posture de dialogue ouvert n'excluant pas Israël et ne l'enfermant pas dans une relation exclusive avec les États-Unis. La France et l'Europe doivent laisser leur porte ouverte à tous les partenaires, et cette logique ne doit pas prendre le pas sur des actes unilatéraux. Poursuivre une logique partisane, c'est l'échec assuré des négociations. La position du groupe Les Républicains est assumée et s'inscrit pleinement dans la politique d'équilibre de la France, héritée du général de Gaulle. Nous appelons à une reprise du processus de négociation dans le cadre du Conseil de sécurité des Nations unies et d'un accompagnement international des Israéliens et des Palestiniens vers la solution à deux États avec une paix complète, juste et durable entre les parties, dans le cadre d'une reconnaissance mutuelle

notre diplomatie est très active au Moyen-Orient pour conclure des accords de coopération militaire, mais un dossier n'avance pas : celui du conflit entre Israël et la Palestine. Cette impuissance est délétère et tragique pour les deux peuples. Pour les Palestiniens, la situation empire : la colonisation de leurs terres s'étend et mite leur territoire. La guerre de Gaza au mois de mai dernier, la quatrième depuis l'instauration du blocus, avec son cortège de morts des deux côtés, de blessés et de destructions, et de destructions, d'engrenage des violences, n'a été suivie d'aucune reprise de pourparlers. Dans une question écrite, je rappelais, comme les organisations internationales, que dans le territoire palestinien occupé, notamment dans la zone C, les besoins fondamentaux de la population civile ne sont plus satisfaits, en termes tant d'infrastructures sanitaires que d'accès aux services essentiels, ce qui est d'autant plus grave en temps de pandémie. En vertu du droit international, les autorités israéliennes sont pourtant tenues de pourvoir aux besoins de la population ou de faciliter les activités humanitaires des tiers. Israël ne remplit pas ces obligations. Pis, les autorités israéliennes dissuadent les bailleurs d'intervenir, entravent l'accès des ONG et continuent de détruire l'assistance humanitaire, y compris celle qui est financée par la France La récente classification par le gouvernement israélien de six ONG palestiniennes de défense des droits, comme organisations « terroristes » et leur interdiction marque une étape supplémentaire dans la répression. Là encore, nous alertons en vain : le Gouvernement proteste, et puis rien L'Union européenne estime que 48 % de la population palestinienne totale a besoin d'une aide humanitaire. Dans la bande de Gaza, ce ne sont pas moins de 80 % des Gazaouis qui ne survivent que par l'action humanitaire. La France a longtemps joué un rôle important dans les négociations pour la paix, et notre action diplomatique ne peut pas se réduire à émettre régulièrement des condamnations impuissantes. En 2014, quelques mois après la troisième guerre de Gaza, et sur la base des résolutions de l'ONU, notre parlement adoptait une résolution appelant à la reconnaissance de l'État de Palestine. Mais, depuis, la situation s'enfonce toujours plus dans l'impasse. Cela nous appelle à reprendre l'initiative

Après trois ans de gel des négociations entre les deux parties, soixante-dix pays avaient réitéré leur engagement pour un règlement pacifique et multilatéral du conflit. L'investiture de Donald Trump a stoppé cette dynamique. Le plan états-unien est allé contre les résolutions successives de l'ONU, légalisant, voire encourageant la multiplication des colonies israéliennes en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, prévoyant l'annexion d'une grande partie de la vallée du Jourdain. L'attachement du peuple palestinien à sa terre est systématiquement attaqué. Au mois d'octobre, les agressions au moment de la récolte des olives des olives se sont multipliées. Selon les Nations unies, quelque 1 300 arbres ont été détruits par les colons. Au premier semestre, l'armée elle-même a dénombré des centaines d'incidents arrachages d'arbres, terres usurpées, dispersion des populations, qui alimentent le cycle de la violence et éloignent la perspective d'une solution politique juste et durable. Aujourd'hui, la population palestinienne s'engage pour la défense de ses droits civiques. À la suite des violences du printemps, une résolution de l'ONU a permis aux enquêteurs de constater l'augmentation importante des actes de violence de la part de colons israéliens contre des Palestiniens.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme le disait mon collègue Pierre Laurent, nous sommes à un tournant historique du conflit israélo-palestinien. Parvenir, dans le cadre d'une initiative internationale, à concrétiser une solution à deux États, qui reconnaîtrait un État palestinien et un État d'Israël, constitue notre seule chance d'aboutir à une paix juste et durable entre les deux peuples.

en moins de vingt ans, sans compter les centaines de millions d'euros de taxes douanières retenus illégalement par Israël. Ce frein au développement est la raison majeure du désastre humain que constitue la colonisation 48 % des Palestiniens et 80 % des Gazaouis ont besoin d'une aide alimentaire pour survivre ; 900 000 Palestiniens souffrent d'un accès limité à l'eau, aux soins, à l'éducation et aux autres services de base. l'accélération de la colonisation et des violences dans les territoires occupés les privent de plus en plus souvent d'un toit. Mais la solution à deux États serait également bénéfique pour les Israéliens, bien que ce point ne soit pas souvent évoqué. En 1988, à Alger, puis devant l'Organisation des Nations unies, Yasser Arafat, alors président de l'Organisation de libération de la Palestine, déclarait : « Notre conseil national palestinien redit son rejet du terrorisme sous toutes ses formes, compris le terrorisme d'État. Notre position est claire et sans ambiguïté. » Alors que 70 % de la population palestinienne a moins de 30 ans, comment penser que les actes de violence qu'elle subit au quotidien n'alimentent pas les tirs de roquette ? Reconnaître l'État de Palestine dans ses frontières de 1967 assécherait ainsi la plus grande partie du vivier de recrutement du Hamas. Se pose par ailleurs la question de la stabilité dans la société israélienne elle-même. Comment comprendre que, en l'espace de deux ans, la Knesset ait adopté une loi sur l'État-nation reconnaissant le caractère juif de l'État, tout en autorisant des colonisations et des annexions qui conduisent à ce que 40 % de la population israélienne soit arabe et palestinienne Revendiquer une solution à deux États ne relève ni de la haine envers l'un des deux peuples, ni du dogmatisme ou de la posture. Cela relève d'une aspiration à la coexistence pacifique de deux États et de deux peuples, ainsi que d'un strict respect du droit international, constant depuis 1947. Cela implique de reconnaître l'existence d'un État arabe palestinien et d'un État juif israélien, mais aussi le droit au retour des réfugiés palestiniens sur des terres qu'ils ont occupées depuis des générations, de reconnaître l'internationalisation de Jérusalem et la cogestion des lieux de culte dans reconnaître les frontières de 1967 dessinées par l'accord d'armistice de 1949, de reconnaître l'illégalité de l'occupation et de la colonisation par Israël de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie, du plateau du Golan et de la vallée du Jourdain,

Cela consisterait simplement à faire preuve de cohérence avec les résolutions de nos instances multilatérales. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, ayant appris des limites de la Société des Nations, nos prédécesseurs ont créé l'ONU, fondée sur le triptyque droit international, objectif de paix et moyens d'action dédiés à la préservation de ladite paix. Le fonctionnement des Nations unies, très certainement à revoir, doit être un point d'appui pour une initiative internationale. La France, présidente du Conseil de l'Union européenne et membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, doit être l'un des moteurs des négociations. C'est pourquoi notre groupe a fait le choix de demander le vote du Sénat sur cette proposition de résolution, que je vous encourage également à soutenir, mes

La proposition de résolution souligne également l'occasion offerte par la présidence française du Conseil de l'Union européenne à partir du 1 janvier 2022. Ce calendrier est évidemment favorable. Nul ne peut, là encore, le contester.

Est-il possible de relancer une initiative internationale en vue d'aboutir à une solution à deux États sur la base d'imprécations et d'anathèmes ? Je ne le crois pas non plus. Mes Mes chers collègues, le texte qui nous est soumis accuse l'État d'Israël « d'aggraver les atteintes aux droits des Palestiniens ». Il le fustige en outre, en rappelant les « multiples condamnations internationales dont a fait l'objet l'État d'Israël, notamment au sujet de la colonisation et de l'occupation des territoires palestiniens ». Enfin, les auteurs de la proposition de résolution jugent « malvenu et déséquilibré le " plan de paix " imposé bilatéralement par les États-Unis d'Amérique et l'État d'Israël en janvier 2020 ». Le plan Trump n'est sans doute pas parfait, mais il trace un chemin pour la paix. Il ouvre la voie à une solution à deux États. Le plan pose une condition légitime : que les dirigeants palestiniens reconnaissent Israël comme un État juif. Il propose une solution pour Jérusalem : la ville serait entièrement sous contrôle israélien, mais la capitale de la Palestine se situerait dans la section de Jérusalem-Est. Elle pourrait éventuellement être nommée Al-Quds, nom de la ville de Jérusalem en arabe. Les deux capitales devraient être internationalement reconnues. Ce sont des propositions raisonnables, qui ne méritent pas d'être balayées d'un revers de main au motif qu'elles seraient « malvenues et déséquilibrées ». Ce plan est également intéressant en ce sens qu'il comporte des mesures garantissant la sécurité d'Israël, sécurité à laquelle nous sommes toutes et tous attachés dans cet hémicycle pour la stabilité du Proche-Orient. Ainsi, l'État de Palestine serait démilitarisé. Il mettrait en place des forces de sécurité pour sa sécurité intérieure et pour empêcher les attentats terroristes en Palestine, en Israël, en Jordanie et en Égypte. L'État de Palestine renoncerait également au contrôle de ses frontières et de son espace aérien. En retour, les Palestiniens auraient accès à des facilités dans les ports israéliens. Mes chers collègues, au sein du groupe d'amitié France-Israël, présidé par notre collègue Roger Karoutchi, nous oeuvrons pour la paix au Proche-Orient. Nous avons d'ailleurs rencontré, le 27 septembre dernier, Émilie Moatti, la nouvelle présidente du groupe d'amitié Israël-France à la Knesset. Elle est par ailleurs vice-présidente de la Knesset et présidente de la sous-commission des affaires étrangères. À notre niveau, nous essayons de rapprocher les points de vue et de favoriser le dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Nous ne pensons pas qu'une telle résolution manichéenne soit de nature à apaiser la situation. Dans une tribune que j'ai cosignée dans en 2014, j'ai dit être favorable, comme de nombreux responsables politiques, à une résolution négociée du conflit israélo-palestinien fondée sur la coexistence pacifique et la reconnaissance mutuelle de deux États vivant en paix et en sécurité. Nous sommes convaincus qu'il n'y a pas d'autre solution que la négociation et que seule la voie du dialogue permettra aux Israéliens et aux Palestiniens d'avancer sur le chemin escarpé de la paix. Le texte proposé rompt de manière inopportune avec la position constante de notre pays, qui oeuvre depuis plus de trente ans en faveur d'une paix fondée sur le principe des deux États, au terme d'un processus de négociation, qui implique de part et d'autre des concessions. Frappée au coin du bon sens, cette ligne diplomatique a fait l'objet d'un large consensus politique au-delà des clivages partisans. Elle repose sur un nécessaire équilibre entre les exigences et les préoccupations de nos amis israéliens et palestiniens.

Vous étiez vingt et cent, vous étiez des milliers Nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés Qui déchiriez la nuit de vos ongles battants Vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent » J'ai souhaité

successives, de part et d'autre des frontières de 1967. C'est pourquoi tous ceux qui souhaitent oeuvrer pour la paix se doivent de répondre à une exigence d'impartialité et de veiller à ne pas envoyer des signaux ou des non-dits qui empêchent les plaies de cicatriser. Sur ce point, mes chers collègues, je regrette la rédaction de votre proposition de résolution,

dont Israël a fait l'objet. Mais il manque un rappel aussi essentiel qu'évident : la condamnation des actes de terrorisme, en particulier ceux qui ont été commis du côté palestinien. Cette lacune entraîne un déséquilibre qui dessert le texte et le détourne de son objectif. Enfin, le dernier considérant invite le Gouvernement, à la veille de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, à relancer une initiative internationale.

Il faut soutenir cette démarche. Sans implication durable et respectée des acteurs de la région, rien ne sera possible. Contrairement à d'autres puissances, la France mobilise, réunit, fédère. ce n'est pas l'esprit du texte proposé. Enfin, mes chers collègues, malgré le contexte géopolitique pour le moins tendu dans tout le Moyen-Orient, je veux croire et regarder vers l'avenir. Nous devons laisser une chance à tous les acteurs

commencer mon propos en rappelant trois évidences. Premièrement, la France est et restera toujours l'amie du peuple palestinien comme l'amie du peuple israélien.

au Proche-Orient. D'ailleurs, l'escalade de violences à Jérusalem, à Gaza et en Cisjordanie en mai dernier a rappelé que ce conflit n'avait rien perdu de sa centralité. La France n'a ménagé aucun effort pour contribuer à la cessation des hostilités.

Malgré tout, plus de six mois après la fin des hostilités, les défis restent multiples : préserver un cessez-le-feu durable à Gaza, auquel l'Égypte a apporté son soutien, assurer la reconstruction et l'appui humanitaire, prévenir toute mesure unilatérale qui contribuerait à une nouvelle escalade. Au-delà, c'est le rétablissement d'un horizon politique crédible qui reste nécessaire pour permettre aux Palestiniens et aux Israéliens de vivre en paix et en sécurité dans le respect des droits de chacun. Très clairement, sans cet horizon politique crédible, il est à craindre que, les mêmes causes produisant les mêmes effets, les cycles de violences ne se répètent, nourrissant un conflit qui n'a que trop duré. Je souhaite à ce propos rappeler que la position de la France demeure constante sur les conditions d'un règlement politique du conflit israélo-palestinien. Cette position repose sur trois éléments excellemment rappelés par Nicole Duranton. Un cadre, tout d'abord : celui du droit international, fondé sur les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies et les paramètres internationalement internationalement agréés. Un objectif, ensuite : l'établissement de deux États vivant effectivement dans la paix et la sécurité au sein de frontières sûres et reconnues, fondées sur les lignes du 4 juin 1967, avec Jérusalem pour capitale de ces deux États. Une méthode, enfin : la négociation entre les parties et l'absence de décision unilatérale. Comme vous le savez, le soutien de la France à la solution des deux États est indéfectible, pour une raison très simple : il n'y a pas d'alternative viable. C'est la seule solution qui puisse répondre de façon juste et durable aux aspirations des peuples palestinien et israélien. et israélien. Tout plan qui viserait à s'éloigner de cette solution est illusoire, car les aspirations d'un peuple ne peuvent se réaliser durablement au détriment des droits et des aspirations de l'autre. Comme l'avait indiqué le Président de la République devant l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2020, la paix ne pourra se construire sur l'hégémonie ou l'humiliation. L'État palestinien doit pouvoir coexister dans la paix et la sécurité aux côtés de l'État d'Israël.

? Pour oeuvrer à la concrétisation de cette solution à deux États, la mobilisation de la France et de la communauté internationale doit être double : d'une part, il faut une action collective pour garantir

de la France au regard de la poursuite, par le gouvernement du Premier ministre Bennett, de la politique de colonisation et des évictions de familles palestiniennes de Jérusalem-Est. La colonisation sous toutes ses formes est contraire au droit international, et elle porte directement atteinte à la solution des deux États. Les risques sont d'autant plus importants que celle-ci est menée dans des zones sensibles pour la contiguïté d'un futur État palestinien. On pense notamment aux zones E1, Givat Hamatos ou Har Homa. Je rappelle à cet égard notre condamnation des annonces faites par les autorités israéliennes à la fin du mois d'octobre de la construction de plus de 4 000 logements en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Notre mobilisation et notre vigilance restent entières, conjointement avec nos partenaires européens. Je tiens également à rappeler la pleine mobilisation de la France l'an dernier pour prévenir l'annexion partielle de la Cisjordanie, qui, souvenez-vous, avait été envisagée par le gouvernement Netanyahu. Nous avions alors clairement affirmé qu'une telle annexion, quel que fût son périmètre, aurait rendu impossible la solution des deux États et mis un terme de façon irréversible à la perspective de création d'un État palestinien viable. La France a été particulièrement active pour envoyer des messages fermes et dissuasifs à cet égard. Ensuite, pour concrétiser la solution des deux États, il faut naturellement préserver la possibilité d'établir un futur État palestinien qui soit viable. Cela passe par un soutien aux institutions palestiniennes et un renforcement de la gouvernance démocratique dans ces territoires, où l'on observe des dérives inquiétantes. La France, comme France, comme les années précédentes, apporte une aide budgétaire de 16 millions d'euros à l'Autorité palestinienne pour financer le plan national de développement palestinien et renforcer les institutions palestiniennes. La France soutient également par ailleurs l'UNRWA, qui agit auprès des réfugiés palestiniens,

palestiniennes de défense des droits de l'homme comme organisations terroristes est très préoccupante- l'une d'entre elles avait reçu le prix des droits de l'homme de la République française en 2018. Mais pour revenir au sujet de la gouvernance palestinienne, la France appelle très clairement à des progrès tangibles pour la renforcer. Des institutions démocratiques fortes, fondées sur le respect de l'État de droit, sont indispensables pour un État palestinien viable. Nous avons d'ailleurs déploré, l'été dernier, les arrestations de membres de la société civile palestinienne, et exprimé notre exprimé notre vive préoccupation à la suite du décès de Nizar Banat après son arrestation par les forces de sécurité palestiniennes. Nous rappelons notre attachement au respect de la liberté d'expression et des droits de l'homme, fondement de toute société démocratique. besoin de s'exprimer démocratiquement et, après un report regrettable cette année, il revient à l'autorité palestinienne d'organiser des élections nationales, selon un calendrier rapproché. Il revient également aux autorités israéliennes d'autoriser la tenue du scrutin à Jérusalem-Est. Enfin, oeuvrer à la concrétisation de la solution des deux États passe par une mobilisation de la communauté internationale pour aboutir à la reprise des négociations entre les parties. L'un d'entre vous a évoqué l'année 1991, il y a trente Israéliens et Palestiniens s'engageaient dans leurs premières négociations, après la conférence de Madrid. De Madrid à Taba, en passant par Oslo et Camp David, ces négociations ont- hélas ! -fait place à une frustration d'autant plus forte que la paix semblait alors à portée de main. ans après Madrid, les négociations entre les parties n'ont jamais paru aussi lointaines et la frustration a cédé la place à l'amertume. Le risque est désormais de voir s'éloigner durablement toute perspective de reprise des négociations entre Israéliens et Palestiniens, tant la défiance est grande de part et d'autre. L'absence de perspectives politiques laisse d'ailleurs la place aux accès de violence, comme est venue le rappeler tragiquement l'attaque terroriste du 21 novembre dernier à Jérusalem, que nous avons condamnée avec la plus grande fermeté. L'urgence est bien de créer les conditions d'une reprise des négociations directes entre les parties pour qu'elles renouent le fil du dialogue. C'est ce à quoi s'efforce la France depuis plus d'un an et demi aux côtés de ses partenaires allemand, égyptien et jordanien, dans le cadre du groupe d'Amman ou du format de Munich, établi au début de 2020 sur notre initiative, peu après la présentation du pseudo-plan du président Trump. Ce format rassemble les ministres des affaires étrangères des deux États européens et des deux États arabes engagés sur le dossier israélo-palestinien, l'Égypte et la Jordanie. s'est déjà réuni à quatre reprises, en étroite coordination avec l'Union européenne et les Nations unies. Ses travaux ont permis dans un premier temps de maintenir à l'agenda la perspective de cette solution à deux États, après l'annonce du plan Trump, et d'accompagner une reprise de la coordination qui est aujourd'hui L'objectif est désormais de poursuivre et d'amplifier ces efforts, complémentaires à ceux du Quartet, en vue de rétablir un niveau de confiance suffisant et, à terme, de créer les conditions d'une reprise directe des négociations. Les récents contacts de haut niveau entre Israéliens et Palestiniens ces derniers mois participent de cette dynamique positive que nous encourageons. Ils s'inscrivent dans un contexte de recomposition régionale qui est positif pour la paix et pour la stabilité régionale, permis notamment par la normalisation des relations entre plusieurs États arabes et Israël, que la France a saluée. Le Président de la République s'est d'ailleurs récemment rendu aux Émirats arabes unis et a eu l'occasion de féliciter les autorités émiriennes pour ce grand pas pour la paix et la stabilité dans la région. des affaires étrangères, Yaïr Lapid, en faveur des territoires palestiniens vont également dans le bon sens. Nous les avons saluées, mais force est de constater que cette dynamique demeure fragile, comme l'illustrent les derniers signaux négatifs sur le terrain les violences, les annonces en matière de colonisation, la crise humanitaire structurelle, le blocus israélien imposé à la population de Gaza, qui subit elle-même le contrôle du Hamas. Mesdames, messieurs les sénateurs, cette résolution invite le Gouvernement à engager une initiative internationale ou européenne sur le dossier israélo-palestinien.

nous soutenons les efforts de l'envoyé spécial de l'Union européenne à ce titre. S'agissant de la reconnaissance de l'État palestinien, elle devra intervenir au moment opportun, dans le cadre et le format appropriés, lorsque cette décision sera directement utile à la paix. Nous l'avons toujours dit : cette reconnaissance doit s'inscrire dans le cadre d'un règlement global et définitif du conflit. Nous ne voulons pas d'une reconnaissance symbolique, qui n'aboutirait qu'à un État virtuel. virtuel. Nous engagerons des démarches en ce sens, le moment venu, dans le cadre d'un processus politique crédible, en vue de l'établissement effectif de deux États sur le terrain.